Officiellement, Ankara souhaite établir le long de sa frontière une zone de sécurité en installant au moins 1 million de réfugiés et en construisant, en un temps record, villes et infrastructures. Mais, dans les faits, ce sont à nouveau des milliers de civils qui sont pris dans l'étau d'une guerre civile qui déchire, depuis 2011, ce pays martyr, avec des conséquences humanitaires terribles on parle de près de 160 000 déplacés, d'exactions, de règlements de compte nourris par des haines longuement mûries. L'offensive turque, qui suit le retrait des troupes américaines, s'inscrit dans ce que l'ancien ambassadeur de France en Syrie, Michel Duclos, appelle « la géopolitique des nouveaux autoritaires ». Ou quand la volonté de puissance intérieure et extérieure des dirigeants turcs, russes ou iraniens a fait de la Syrie le terrain de jeu mortifère de leurs ambitions. Ne nous y trompons pas : ce qui se passe met gravement en cause la stabilité régionale et internationale, avec en toile de fond le retour en force de Bachar al-Assad, le spectre de la résurgence de Daech, que les forces kurdes ont combattu, mais qui, comme l'hydre, n'a jamais totalement disparu, la pantomime pathétique d'une OTAN déchirée, le spectacle désolant d'une Europe militairement impuissante- et nous reconnaissons l'engagement du Président de la République en faveur d'une armée européenne. Oui, la France entretient des liens d'amitié profonds et anciens avec le peuple turc Mais le chantage de ses dirigeants est insupportable. Il appelle de notre part la plus grande fermeté. Monsieur le Premier ministre, que va faire la France pour faire cesser l'offensive turque et le drame humanitaire qui s'annonce ? Comment agira-t-elle pour empêcher la fuite des djihadistes français aujourd'hui détenus ? Quelles sont nos marges de manoeuvre pour tenter de stabiliser cette région ?

considérable tant par les moyens qu'elle mobilise, avec le soutien massif de supplétifs syriens de l'armée nationale syrienne,

Le 13 octobre, les États-Unis ont décidé, là encore de manière unilatérale, de retirer leur dispositif militaire du nord-est syrien. Ces deux décisions unilatérales emportent des conséquences très lourdes des conséquences très lourdes pour nos partenaires kurdes, qui se sont battus à nos côtés contre Daech, hommes et femmes réunis, et à qui je veux rendre une nouvelle fois hommage en notre nom à tous.

L'idée que l'État islamique puisse reprendre pied de façon organisée, que ce soit au nord-est syrien ou, le cas échéant, à travers la déstabilisation de la région, au nord-ouest irakien fait peser un risque sécuritaire sur l'ensemble de la région et sur l'ensemble de nos pays pour les raisons que nous n'ignorons pas. Conséquences très lourdes encore sur le plan humanitaire : 700 000 civils se trouvent des familles entières ont pris la route pour fuir les combats. Depuis le début de l'offensive, on dénombre 150 000 déplacés et, bien évidemment, de premières victimes civiles. Conséquences très lourdes, enfin, sur la recherche d'une solution pérenne dans la région : l'offensive militaire et les menaces de la Turquie de réinstaller, de force, les réfugiés syriens en Turquie, dans la zone des trente kilomètres qui longe la frontière entre la Syrie et la Turquie, ne vont pas faciliter l'avènement d'une solution l'avènement d'une solution politique dans la région. Monsieur le président Requier, vous posez la question de la réaction de la France. Nous avons pris un très grand nombre d'initiatives. D'abord, la France a, de la façon la plus claire et la plus ferme, condamné cette opération militaire. Nous l'avons dit à l'ambassadeur de Turquie en France, par l'intermédiaire du Quai d'Orsay. Le Président de la République a eu l'occasion de s'entretenir avec le Président Erdogan : il lui a dit clairement quelle était la position de la France et lui a signifié notre condamnation de cette opération militaire. Nous avons ensuite cherché à mobiliser dans les enceintes internationales,

Face à l'impact de cette opération militaire sur la sécurité européenne, nous avons décidé, avec d'autres pays, de suspendre nos exportations d'armes vers la Turquie. C'est une décision commune de l'Allemagne, des Pays-Bas, de la Norvège, de la Finlande et du Royaume-Uni. Le Canada a pris la même décision.

compte tenu des décisions turques et de l'unilatéralisme dont ce pays a fait preuve, ne nous voilons pas la face : demander, condamner, inciter, nous le ferons ; obtenir, ce sera beaucoup plus difficile- ce le sera d'autant

Cette agression est un crime contre la paix, contre les combattants kurdes qui se sont battus contre Daech et contre l'expérience d'un Rojava démocratique. Elle offre une opportunité inespérée à Daech de reconstruire ses forces. Nous avions alerté à de nombreuses reprises sur les risques de voir la Turquie franchir le pas, sur les ambiguïtés de la coalition et sur le rôle trouble joué par la Turquie en son sein. Aujourd'hui, les masques tombent. La Turquie fait la guerre aux Kurdes, et à personne d'autre, au mépris de la sécurité du monde. Et cette guerre a été autorisée par le Président des États-Unis La France doit parler d'une voix claire, forte, indépendante, qui ne s'étouffe pas aussitôt dans les coulisses du renoncement. La France doit agir. Premièrement, au-delà de l'embargo annoncé à quelles sanctions économiques, financières et politiques fortes la France est-elle prête ? La Turquie est un important partenaire commercial, nous avons donc les moyens d'agir. Deuxièmement, la France continue-t-elle d'agir pour aboutir à la mise en place d'une zone d'exclusion aérienne ? Et comment ? Troisièmement, que répond la France à l'appel lancé par quinze organisations humanitaires ? Quelle est notre stratégie pour obtenir un cessez-le-feu qui protège le travail humanitaire, garantisse son accès en tout lieu, qui protège les populations civiles par l'interdiction de l'utilisation des armes explosives en zones peuplées, qui permette de rapatrier les enfants français détenus dans les camps de prisonniers prisonniers ? Enfin, puisque les États-Unis et la Turquie sont au coeur de cette affaire et qu'ils sont membres de l'OTAN, n'est-il pas temps de convoquer un débat parlementaire d'urgence interrogeant le rôle de l'OTAN, notre rôle dans cette alliance et notre place au sein de son commandement intégré ? Le Gouvernement est-il prêt à convoquer d'urgence ce débat parlementaire ?

La France est intervenue activement au sein du Conseil des ministres des affaires étrangères, lundi dernier. C'est parce qu'une voix forte s'y est exprimée, celle de Jean-Yves Le Drian, qu'une condamnation unanime, je crois,

au Président Erdogan. La France continuera à être mobilisée pour obtenir la cessation de l'offensive turque contre les Kurdes le plus rapidement possible. Ce sujet nous engage chaque heure, chaque jour, chaque semaine, tant que cette situation

Il y va de la fidélité à nos alliés kurdes, bien évidemment, et à nos valeurs, mais aussi de notre propre sécurité, comme le Premier ministre l'a lui-même Chacun sait le rôle exceptionnel des combattants kurdes, aux côtés de la coalition internationale, dans l'éradication du califat de Daech. Chacun sait que, les attaquer aujourd'hui, c'est permettre la résurgence du terrorisme islamiste jusque sur notre sol. Le Président de la République a appelé la société française à faire bloc contre le terrorisme.

Cessons d'intérioriser un sentiment d'impuissance et d'isolement largement exagéré. L'invasion par la Turquie du canton d'Afrin, livré ensuite aux milices djihadistes et où les Kurdes ont été victimes d'un véritable nettoyage ethnique, était un avertissement auquel nous n'avons pas su réagir. La France va-t-elle enfin se mobiliser à la hauteur des sacrifices réalisés pour nous par les combattants kurdes ?

Monsieur le sénateur, je vous sais très impliqué sur la question kurde, à l'image de la Haute Assemblée et de sa commission des affaires étrangères, qui, ce matin, a auditionné l'ambassadeur de Turquie. Je veux saluer saluer la proposition de résolution qui appelle à un engagement résolu de la France en faveur de toute initiative. Sachez que nous rejoignons

nous nous préparons d'ores et déjà à une réponse avec notre centre de crise et de soutien. Un afflux de réfugiés risque de se produire au Kurdistan irakien. Une demande d'aide internationale a été formulée pour pouvoir gérer cette situation. Nous devrons être également présents au rendez-vous pour ces frères d'armes dans la lutte contre le terrorisme que sont les Kurdes. les autorités françaises à s'engager davantage et à sortir de la posture défensive dans laquelle nous nous sommes nous-mêmes placés. Rappelons-nous la phrase de Charb Contre le cynisme et la mort, aujourd'hui, il y a le peuple kurde. » Il est de notre devoir et de notre intérêt d'être à ses côtés ; nous serons à vos côtés pour prendre des initiatives beaucoup plus fortes dans les jours qui viennent.

Malgré l'annonce de l'imminence d'un possible accord la nuit dernière entre l'Union européenne et le Royaume-Uni concernant le Brexit, la pression qui pèse sur le Conseil européen de demain

pour l'heure- faut-il le rappeler ? -, le Royaume-Uni fait encore partie de l'Union européenne, et les interrogations quant aux relations futures ne cessent de grandir. Ce fut notamment le cas lorsque, le 3 juin dernier, le Président américain, Donald Trump, tweetait : « Un grand accord commercial est possible une fois que le Royaume-Uni se sera débarrassé de ses chaînes.

d'ailleurs été conclu le 3 octobre dernier, non sans remous. La Commission européenne, saisie de cette question, doit se pencher sur la conformité de tels accords avec le droit communautaire. Beaucoup d'incertitudes demeurent encore, elles sont plus fortes encore pour nos entreprises. Nous entendons les craintes et les inquiétudes de nos concitoyens et de nos PME dans nos territoires. Quelles mesures concrètes comptez-vous mettre en place pour préparer l'après-Brexit, à la fois en termes économiques, mais aussi politiques ? La parole est à M. le

Les préparatifs ont continué à se faire de façon intensive sous la houlette du Premier ministre, qui réunit très régulièrement tous les ministères concernés. S'agissant des entreprises, dont vous évoquez les inquiétudes, nous avons conduit une action très proactive à leur égard, y compris en appelant individuellement chacune des entreprises exportatrices françaises vers le Royaume-Uni, pour préparer toutes les procédures en cas de non-accord. des heures et jours prochains, un éventuel accord aboutir ? Michel Barnier a estimé la semaine dernière que des garanties suffisantes existaient pour une reprise pleine et entière des négociations, mais l'heure tourne

L'Union européenne se montre clairement ouverte à la négociation. Elle est constructive dans les discussions. Mais encore faut-il que le Premier ministre britannique donne l'impulsion politique nécessaire. Son cabinet doit se réunir dans les prochaines heures, nous dit-on. Quelle que soit l'évolution, nous sommes prêts à faire face à tous les scénarios, y compris à celui d'un retrait sans accord. Nous avons adopté des cadres juridiques très complets, la sensibilisation a été conduite, et nous avons organisé une coordination très active avec tous les pays voisins. Au-delà du 31 octobre prochain, tout restera à faire pour bâtir une relation future. L'histoire est là, la géographie est là : le Royaume-Uni reste un pays européen, au sens large du terme, et nous devrons bâtir une relation qui reste proche, compte tenu de ces liens. La parole

déjà près de 1 000 morts à l'heure où nous parlons, 160 000 civils jetés sur les routes, le retour de Daech et le risque, peut-être pire encore, d'évasion de djihadistes, qui viendront faire payer très cher à l'Europe son engagement. Enfin, les Kurdes, les Kurdes, nos alliés, nos amis, qui se sont battus avec tant d'héroïsme pour notre propre sécurité, ce peuple sans patrie, trahi une fois de plus, sont contraints d'appeler au secours leurs ennemis d'hier. Les Américains ont cru défendre leurs intérêts, mais quelle confiance accordera-t-on demain à leur parole ? Monsieur le Premier ministre, mes questions sont simples : comment l'OTAN peut-elle rester sans réagir ? Nous étions un certain nombre dimanche dernier à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. À nos questions, fortes- nous avons fait entendre la voix de la France -, le secrétaire général Stoltenberg n'a jamais daigné répondre. Par ailleurs, que comptez-vous faire face aux milliers de djihadistes qui menacent notre sécurité ?

Si le principe d'une alliance est de permettre à des partenaires de travailler ensemble, les décisions unilatérales ou celles qui s'entrechoquent les unes avec les autres ne me paraissent pas relever d'un bon fonctionnement.

façons. Tout d'abord, il y a la reconstitution d'un espace géographique maîtrisé par Daech, lequel serait propice à l'organisation d'actions à l'extérieur de ce territoire.

évidemment prêts à judiciariser tous ceux qui, s'étant rendus sur zone, se sont rendus complices des actions criminelles qui ont été conduites sur place.

aux prescriptions du préambule de la Constitution de 1946, aux termes duquel « l'organisation de l'enseignement public gratuit à tous les degrés est un devoir de l'État ». Seuls des tarifs modiques seraient autorisés. Le jugement répond à une question prioritaire de constitutionnalité sur la possibilité donnée aux universités d'augmenter significativement les droits d'inscription pour les étudiants étrangers, la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat avait demandé un moratoire. Cependant, la portée de cette décision dépasse la simple question des tarifs appliqués aux étudiants étrangers et s'applique aux droits d'inscription de l'ensemble des étudiants, français et étrangers, dans l'ensemble des établissements publics, universités Ce jugement, que le Conseil constitutionnel qualifie lui-même d'inédit, crée des incertitudes juridiques, tant il est difficile à ce jour d'en mesurer toutes les conséquences. Il pose un certain nombre de questions qui pourraient avoir un impact sérieux sur le financement de nos établissements. Le principe d'autonomie financière n'est-il pas atteint par cette décision, qui remet en cause la possibilité pour les établissements de fixer eux-mêmes leurs droits d'inscription ? La gratuité est-elle réellement un moyen efficace

Enfin, monsieur le ministre, pouvez-vous partager avec nous la lecture que fait le Gouvernement de ce jugement ? Quel en sera l'impact sur le financement des établissements de l'enseignement supérieur ? Quelles conséquences entraîne-t-il sur la hausse des frais universitaires pour les étudiants étrangers, décidée dans le cadre du plan Bienvenue en France ?

Mme la ministre de l'enseignement supérieur, Frédérique Vidal, qui est actuellement aux côtés du Président de la République au conseil des ministres franco-allemand. Vous l'avez rappelé, une question prioritaire de constitutionnalité a été déposée auprès du Conseil constitutionnel à la suite de l'examen d'une requête par le Conseil d'État.

Le Conseil a également rappelé que le financement de l'enseignement supérieur devait principalement- mais pas exclusivement -être assuré par l'impôt et qu'il convenait de prendre en compte la situation financière de chaque étudiant. Le ministère a pris acte de cette décision. Désormais, il reviendra au Conseil d'État de statuer ultérieurement sur le fond de ce litige. Vous le savez, le plan Bienvenue en France et, de façon plus générale, les enjeux de financement de l'enseignement supérieur font l'objet d'une réflexion collective, dont vous avez rappelé certains tenants et aboutissants. le plan Bienvenue en France, la commission de la culture a étudié le sujet en détail voilà quelques mois. Il s'agit de nous donner les moyens d'accueillir mieux un plus grand nombre d'étudiants internationaux.

Chacun pourra le constater, les deux critères dégagés par le Conseil constitutionnel, à savoir la prise en compte des situations individuelles et le financement à titre principal par l'impôt, sont respectés, ce qui peut nous rendre optimistes pour la suite.

Le Conseil d'État tranchera dans les prochains mois. Sa décision répondra définitivement aux interrogations qui demeurent à ce stade. La parole est à M. Julien Bargeton, pour le groupe La République En Marche.

qui a été présenté hier par plusieurs ministres. Il doit fonder un économique, écologique et technologique. L'industrie française dispose d'atouts,

Des emplois industriels se créent, mais des sites sont menacés. Le mérite de ce pacte est de ne pas minimiser les enjeux auxquels nous devons faire face pour répondre à la demande mondiale. Certains secteurs clés doivent devenir exportateurs nets. Quels sont, selon vous, les leviers principaux pour renforcer notre industrie ? Ont été évoqués, notamment, les impôts de production,

Comment l'industrie peut-elle participer au retour au plein emploi à l'horizon de 2025 ? Ce n'est pas une utopie ! En effet, ce sont les salariés qui rendent possible une nation productive. Quelles sont les actions prioritaires, la méthode envisagée et selon quel calendrier ? La parole

C'est particulièrement vrai dans l'industrie, puisque- je suis heureux que votre assemblée le salue -, pour la première fois depuis dix ans, l'investissement est au plus haut et, pour la première fois depuis dix ans, mesdames, messieurs les sénateurs,

Les Républicains. Ma question s'adresse à M. le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, je souhaite vous interroger à partir de mon expérience, celle d'une élue qui a vu progresser dans nos quartiers le communautarisme, qui a vu les jeunes femmes se mettre à porter le voile sous la pression, alors que leurs mères s'en étaient libérées. Le voile, en 2019, n'est pas anodin, et nous aurions tort de considérer que l'expression d'une pratique religieuse. D'ailleurs, beaucoup de femmes musulmanes, dans notre pays, ne le portent pas. Le voile est trop souvent le symbole d'un islam politique, qui considère la femme comme un « objet soumis » plus que comme un « individu un « individu émancipé », pour reprendre un qualificatif cher au Président de la République. Nous aurions tort de baisser les yeux et de ne pas voir que le port de signes religieux ostentatoires dans le cadre des sorties scolaires est un instrument de prosélytisme et parfois même de provocation. L'école de la République doit montrer aux petites filles qu'elle ne transige pas avec les principes de laïcité et d'égalité. Or, sur cette question centrale du respect de la laïcité et de la neutralité religieuse des adultes intervenant dans le cadre de l'école hors les murs, la majorité et le Gouvernement se divisent. Vous avez tenté, monsieur le Premier ministre, de désamorcer les querelles au sein de votre majorité, mais, une fois de plus, vous avez, en définitive, baissé les bras. Vous ne cessez de dire qu'il faut lutter contre le communautarisme et, en même temps, vous ne cessez de renoncer à agir. Ce n'est pas l'ambiguïté qui contribuera au réarmement moral de notre pays et au respect des principes qui font la France et qui unissent les Français. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous dire exactement ce que le Gouvernement compte faire vraiment pour lutter contre la communautarisation de notre société et faire respecter les principes de notre République laïque et indivisible

d'autant plus qu'il est un outil pour le XXI siècle. La laïcité est on ne peut plus moderne ; elle nous est très utile : dans la société d'aujourd'hui, en effet, nous avons besoin d'une République une, de citoyens égaux. Ce point est très important- c'est ce qui nous différencie d'autres pays, y compris de pays voisins. anglaise, par exemple, est une société communautariste, avec les dangers que cela représente. Oui, vous avez raison, donc : la République et la laïcité sont nos outils d'organisation.

il y a la lutte contre le communautarisme, ce dont je viens de parler : l'enjeu républicain d'une société de citoyens égaux veillant en particulier à l'égalité entre les hommes et les femmes. Enfin, il y a la laïcité, qui s'applique évidemment à toutes les religions et qui est notre bien précieux, parce qu'elle nous permet à tous de vivre ensemble. L'école est la matrice de cette laïcité,

nous ne souhaitons pas une loi, parce qu'une loi créerait plus de problèmes que de solutions : elle serait contre-productive, y compris eu égard à l'enjeu républicain qui consiste à scolariser tous les enfants et à faire en sorte que tous les parents se sentent bienvenus à l'école de la République.

n'ai rien entendu de très concret, mais je ne peux pas croire que, aujourd'hui, vous puissiez rater une occasion de faire montre d'une réelle volonté de lutter contre les velléités de l'islamisme en France, alors que deux Français sur trois sont prêts à soutenir la proposition de loi interdisant le port du voile pendant les sorties scolaires. Franchement, je trouve qu'il y a là un manque de courage

dernier, en séance du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, le président d'un groupe qui n'a rien de républicain a fait dégénérer les échanges, en accusant d'abord les agents de la région d'être touchés par la radicalisation et le communautarisme islamiste, en tweetant ensuite sur la perte d'appétit que provoque chez lui une exposition consacrée à Martin Luther King, en agressant verbalement, enfin, une femme voilée. Des enfants venus découvrir les institutions républicaines sont repartis dans le tumulte et une maman accompagnatrice sous la menace « de l'arrivée des Russes ». Allons ! Certains ont vu dans ces événements une interrogation sur la laïcité. J'y vois surtout la triste expression du racisme. Que nous croyions au ciel ou que nous n'y croyions pas, nous avons la responsabilité de dénoncer le climat malsain qui règne dans ce pays. Les musulmans, pour ce qu'ils sont, sont pointés du doigt. M. Zemmour, récemment condamné, a son rond de serviette sur les plateaux de télévision. Dans les universités, des fichages tendancieux commencent à apparaître. Nous ne tomberons pas dans les pièges tendus par les provocateurs de tous bords. Vous y tombez tout seuls ! Notre boussole, c'est la concorde républicaine. Le Président Macron et vous-même, monsieur le Premier ministre, avez rappelé l'état du droit en ce qui concerne la laïcité.

se passionnent et se divisent autour d'une question, en l'occurrence celle du voile. Je ne méconnais en rien l'importance de ce sujet,

extrêmement exigeants, celui de la neutralité absolue des pouvoirs publics et des agents publics et celui de la liberté de nos concitoyens à croire ou à ne pas croire et à exercer leur culte dans le respect de la loi. Ces principes

en l'occurrence du voile, dans les enceintes scolaires : à l'école, au collège et au lycée. Cette loi a été jugée constitutionnelle. C'est donc un principe qui nous oblige. Mais cette loi n'a pas dit

le Parlement aura vocation à en débattre. La boussole ayant été définie- c'est le droit tel qu'il est aujourd'hui -, le cap me semble devoir être celui de la lutte contre la radicalisation et contre le communautarisme.

proposition de loi portée par Mme la sénatrice Gatel, d'exercer un contrôle beaucoup plus strict sur les écoles hors contrat au moment de leur création ; faire en sorte aussi, grâce à la loi portée par M. le ministre de l'éducation nationale, d'exercer un contrôle beaucoup plus strict sur les enfants déscolarisés, sur les raisons de leur déscolarisation et sur le contenu de l'éducation qu'ils reçoivent à domicile. Voilà des sujets bien plus importants, bien plus porteurs, que ne l'est la proposition de loi qui a été évoquée ! Voici ma position lutte contre la radicalisation, lutte politique contre le communautarisme, lutte à tous les instants, soutien aux enseignants, création des instruments nécessaires. Telle est la position du Gouvernement, la boussole que nous avons choisie, le cap que nous suivons le Premier ministre ; il y a aussi une forme de racisme, qu'il faut dissiper. Des vents mauvais soufflent sur notre société. Il faut dissiper la confusion, apaiser les tensions et ramener tous nos concitoyens vers la République.

qui ne sont plus leur coeur de métier, avec une forte augmentation des incendies, ils joignent leurs revendications à celles des personnels des hôpitaux, eux-mêmes débordés par l'explosion de l'ensemble des services hospitaliers, notamment des urgences. Toutes les professions au coeur des grandes missions de l'État sont en crise profonde. Les policiers vous ont exprimé récemment leur colère ; le suicide récent d'une directrice d'école, la tentative de suicide d'une principale montrent que l'éducation nationale n'est pas épargnée. Cette colère généralisée exprime avant tout une crise de l'autorité de l'État, vertu capitale pour une société. Ces professions qui enseignent, qui soignent, qui nous protègent en ont assez des grands discours qui ponctuent une situation en incessante dégradation, assez de leurs conditions de travail, assez de la violence croissante dont ils sont victimes parce qu'ils représentent l'État. Lorsque l'on touche à un pompier ou à un enseignant, lorsque l'on insulte un médecin, c'est la République que l'on défie. Cette année, 1 272 agressions de pompiers ont déjà été recensées, et 312 pompiers ont été blessés. Nous avons le sentiment que vous assistez en spectateur à une situation qui vous échappe. Pourtant, c'est bien une décomposition de l'État républicain qui se produit sous nos yeux- les événements d'hier en témoignent parfaitement. L'État régalien n'assure plus sereinement, ses grandes missions de service public. Comptez-vous, monsieur le Premier ministre, répondre à la colère et aux angoisses des agents qui rendent service au public ? Qu'avez-vous à dire aux pompiers, aux personnels soignants, aux enseignants, aux policiers, dont la situation se dégrade de manière accélérée ?

Vous avez évoqué la question importante des agressions dont sont victimes les sapeurs-pompiers, souvent du fait même des personnes qu'ils vont secourir, parce qu'elles ont des difficultés psychologiques ou sont sous l'emprise de l'alcool. Il existe bien une montée des violences ; nous la prenons en compte, dans le cadre de conventions de coordination passées avec les policiers

est menée dans le cadre d'une grande concertation avec les organisations syndicales de sapeurs-pompiers. Celles-ci ont été reçues par le ministre de l'intérieur en marge du congrès de Vannes, puis, hier, au cabinet du ministre. Nous allons poursuivre cette discussion

madame la sénatrice, que ce gouvernement met tout en oeuvre pour que l'action des services régaliens, qu'il s'agisse, évidemment, de la sécurité civile, des sapeurs-pompiers, mais aussi de nos policiers et de nos gendarmes, s'effectue dans les meilleures conditions possible. Je pense aux efforts que nous faisons en matière de recrutement,

Union Centriste. Ma question s'adresse à M. le ministre de l'intérieur. Elle est aux confins de deux sujets que nous avons déjà évoqués : le Brexit et le terrorisme. Le Brexit, avec ou sans accord, se traduira par un recul significatif de la coopération policière et judiciaire entre les pays de l'Union européenne et la Grande-Bretagne et par une fragilisation de l'acquis des leviers d'action que nous avions mis en place ces dernières années au service de notre sécurité. est ainsi créée dans la sécurité européenne, d'autant que le Royaume-Uni est l'un des pays les plus touchés par le terrorisme. Il est le deuxième pays occidental, après la France, s'agissant du phénomène des filières syriennes, qui revient au coeur de l'actualité. Le Royaume-Uni ne pourra plus utiliser le système d'information Schengen, qui permet notamment d'alerter sur les déplacements. Fini également l'accès au PNR, au système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages ou à la base de données qui répertorie les empreintes digitales de tous les demandeurs d'asile

Actuellement, les mères de famille valident huit trimestres dans le secteur privé par enfant né ou adopté et quatre trimestres dans le public. C'est ce qu'on appelle la majoration de durée d'assurance. La réforme envisagée vise à supprimer les dispositifs actuels pour les remplacer par une majoration retraite de 5 % par enfant dès le premier enfant. Cette bonification pourra éventuellement être transférée au père ou partagée avec lui. La retraite des femmes est actuellement inférieure de 38 % à celle des hommes. C'est en grande partie dû à la maternité, qui conduit un grand nombre de femmes à prendre du temps pour leur enfant, à renoncer à une promotion, à prendre un temps partiel ou un congé parental. Pour beaucoup de mères n'ayant pas des carrières complètes, l'attribution d'une retraite qui soit le strict reflet de leurs périodes d'activité sera défavorable par rapport au système actuel. Il est particulièrement injuste de bonifier la retraite d'un parent en pourcentage, en lésant les mères dont les carrières sont incomplètes, mais aussi celles ayant de petits salaires. Il serait particulièrement inéquitable que la réforme des retraites accroisse l'écart de niveau de retraites au détriment des mères. Monsieur le haut-commissaire, cette majoration de 5 % se substituera-t-elle à la majoration de durée d'assurance, pénalisant ainsi les femmes ayant élevé plusieurs enfants ? Par ailleurs, cette loi aura-t-elle un effet rétroactif en supprimant les droits acquis par les femmes ayant eu des enfants avant l'entrée en vigueur de la réforme en 2025 ?

Notre cap est clair : les mêmes règles pour tous, l'universalité et la recherche de l'équité. Vous l'avez souligné, quand vous êtes maman dans le secteur public ou dans le secteur privé, vous ne bénéficiez pas de la même majoration de durée. C'est

Le dispositif a été créé pour compenser les préjudices de carrière. Vous l'avez souligné à juste titre, l'Insee, en 2019, a indiqué qu'il existait une perte de 25 % des revenus salariaux des femmes.

deux tiers des hommes ! Nous avons décidé de compenser ce phénomène par une majoration proportionnelle dès le premier enfant, de façon à ce que l'écart de 40 des pensions entre les hommes et les femmes, qui tombe à 25 % avec la réversion, puisse, dans nos simulations, sur les générations 80-90, augmenter les pensions en moyenne des femmes de 5 % à 10 %.

euros, ce qui apportera une amélioration pour les femmes, notamment celles à temps partiel. Le Conseil d'orientation des retraites a indiqué que le dispositif que nous mettions en place était favorable aux carrières heurtées et courtes. Il concerne donc, notamment, les femmes. Voyez-vous, nous avons la prétention d'aller vers davantage de redistribution en faveur des femmes dans le système universel

des outre-mer. En Guadeloupe, en Martinique et en Guyane, le journal ou appartient à un groupe de presse en cessation de paiement. L'unique quotidien régional sera bientôt, peut-être dans un mois et demi, en liquidation. Ces territoires doivent pouvoir conserver une presse vivante et pluraliste, une presse qui a contribué au développement de la citoyenneté, de la liberté d'opinion et de la démocratie dans nos îles. Les mutations technologiques des réseaux sociaux et les changements dans les habitudes de consommation mettent cependant en cause la survie de ce journal. Sa disparition signifierait la perte cumulée de deux cent cinquante-trois emplois à haut niveau de qualification en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane. Ces emplois sont occupés en grande partie par des originaires. Leur niveau de spécialisation rendra leur réembauche difficile, voire impossible en cas de liquidation. Ce quotidien est aujourd'hui constitutif du patrimoine de ces territoires. Depuis plus de cinquante-trois ans, il rythme notre vie quotidienne, il doit être à ce titre préservé. C'est pourquoi il est nécessaire de mobiliser l'ensemble des aides au pluralisme de la presse périodique régionale. Le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État ont consacré, dans leur jurisprudence, la valeur constitutionnelle du pluralisme de la presse écrite. Ils ont également admis qu'un soutien public accru devrait être apporté à la presse d'information politique et générale. Je vous prie, madame la ministre, de nous faire connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre pour maintenir une presse quotidienne régionale vivante, ainsi que les nombreux emplois, si importants pour des territoires touchés par un chômage de masse qui en dépendent.

Le groupe France-Antilles a été placé en redressement judiciaire le 25 juin. Le tribunal de commerce de Fort-de-France se prononcera à la fin du mois de novembre. Des offres de reprise sont d'ores et déjà déposées. Le Gouvernement est mobilisé depuis quelques mois sur ce sujet et a pris trois décisions.

des outre-mer, le comité interministériel de restructuration industrielle, le CIRI, qui a pour mission d'aider les entreprises en difficulté avec des solutions définies entre actionnaires et créanciers,

Comme vous l'avez souligné, le dynamisme d'une presse régionale est fondamental dans nos territoires d'outre-mer comme partout. C'est le droit à l'information, et c'est bien sûr aussi la vie démocratique qu'il nous faut défendre

Le 10 octobre dernier, le groupe Michelin, fleuron industriel français, leader mondial du pneumatique, a annoncé la fermeture définitive du site de La Roche-sur-Yon. Après Joué-lès-Tours en 2013 et 730 emplois supprimés, cette décision met fin à la production de pneus destinés aux poids lourds en France. hommes et femmes hautement qualifiés sont concernés et vont perdre leur emploi. La moyenne d'âge des salariés est de trente-neuf ans, et beaucoup ont été recrutés ces cinq dernières années dans le cadre du plan Skipper, qui prévoyait 100 millions d'euros d'investissement et 200 recrutements. 70 millions qui ont été investis. Des femmes et des hommes ont consenti beaucoup d'efforts pour améliorer la productivité du site. Cela n'a apparemment pas suffi, et le couperet est tombé brutalement. Michelin propose 120 millions d'euros pour accompagner la reconversion de l'usine, suggère la mobilité interne pour des personnes qui ont construit leur vie familiale et professionnelle en Vendée, pour certains depuis plus de trente ans. C'est une vue de l'esprit La présidente de la région Pays de la Loire, Christelle Morançais, et Bruno Retailleau ont obtenu le remboursement des aides régionales accordées à Michelin. Est-ce que l'État fera la même démarche pour une part du CICE ? L'État sera-t-il présent aux côtés des salariés et des élus locaux, dont le maire de La Roche-sur-Yon, Luc Bouard, et le président du département, Yves Auvinet, pour obtenir toutes les garanties et amortir les conséquences de ce drame économique et humain à long terme ? Cette malheureuse actualité illustre les travers de notre économie. Plus généralement, comment l'État entend-il oeuvrer pour préserver et développer l'industrie dans notre pays

Le site de La Roche-sur-Yon est un bassin d'emplois industriels dynamique. J'ai eu l'occasion, quand j'étais dans l'industrie, de travailler sur le sujet. Il faut donc que chaque salarié retrouve un emploi dans les semaines et les mois à venir. Le Gouvernement y sera très attentif.

se vendent mieux et évincent des technologies françaises plus durables et plus écologiques. C'est également un sujet sur lequel le Gouvernement souhaite se mobiliser. Bruno Le Maire et Agnès Pannier-Runacher ont demandé un contrôle express à la DGCCRF. Nous voulons porter ce débat au niveau européen pour faire respecter

l'exigence constitutionnelle selon laquelle « la gratuité s'applique à l'enseignement supérieur public ». Des frais d'inscription « modiques » peuvent néanmoins être perçus, en tenant compte des « capacités financières des étudiants À travers cette décision, qui fait suite à la volonté du Gouvernement d'augmenter brutalement et de manière importante les droits d'inscription pour les étudiants extracommunautaires, il est rappelé que l'égal accès devant l'instruction, aux fondements du projet émancipateur de la République, ne s'arrête pas aux portes de l'enseignement supérieur public et que ce principe ne peut être entravé pour des motifs pécuniaires. Dans l'attente de la décision du Conseil d'État, Mme la ministre de l'enseignement supérieur a dit « vouloir garder la stabilité du système d'enseignement supérieur public ». Très bien ! Mais, comme le dit le poète, « être patient, ce n'est pas attendre, c'est agir en attendant

comment comptez-vous sécuriser et assurer la pérennité du financement de l'enseignement supérieur public, qui risque, on le sait, d'être profondément bouleversé ? La parole est à M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Madame la

C'est votre prisme. Mais la question doit être également examinée au regard de l'exigence de gratuité et d'égalité. Je ne suis pas certaine que payer plus de 2 000 euros de frais d'inscription pour une formation soit une somme modique somme modique pour les étudiants et leur famille. Eh oui ! Nous souhaitons un vrai débat parlementaire, car il s'agit de l'enjeu et du financement de notre enseignement supérieur public demain.

s'adresse à M. le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, par le passé, les immigrés qui venaient en France voulaient s'intégrer dans notre société. Aujourd'hui, les flux migratoires sont différents. Ils conduisent à des noyaux communautaristes qui rejettent notre façon de vivre. Or les terroristes musulmans trouvent leur vivier de recrutement dans le communautarisme radicalisé. Cette radicalisation recrute elle-même dans le communautarisme ordinaire. Il est urgent de réagir. J'approuve la ministre des collectivités territoriales, qui suggère d'interdire le port du voile islamique dans les assemblées des collectivités territoriales. J'approuve aussi la position du ministre de l'éducation nationale, qui ne souhaite pas que les parents qui accompagnent les sorties scolaires portent le voile islamique. Cependant, au Gouvernement, d'autres ministres disent le contraire et soutiennent le communautarisme islamique, au risque de favoriser le terrorisme. De son côté, le Président de la République se complaît dans l'ambiguïté. Monsieur le Premier ministre, oui ou non êtes-vous favorable au port du voile islamique dans les assemblées des collectivités territoriales ? Oui ou non êtes-vous favorable au port du voile islamique par les parents qui accompagnent les enfants dans les écoles ?

quels sont les fondements de notre République et la manière dont le fait religieux est encadré dans l'espace de la République française. La loi de 1905, le Premier ministre l'a rappelé, fixe ce cadre et détermine le fait que, en France, c'est l'État qui est laïque et non pas la société. Ce cadre juridique a été complété il y a quelques années, en 2004,

de communautarisme religieux et contre toutes les formes de radicalisation religieuse. Nous sommes, monsieur le sénateur, tout aussi fermes pour dénoncer toutes les stigmatisations à l'intention de nos compatriotes en raison de leur appartenance à une religion, en particulier à la religion musulmane. Nous sommes une nation ouverte, mais une nation ferme

le conseiller régional du Rassemblement national qui a posé le problème mériterait une décoration, car il a raison ! Nous en avons terminé avec les questions d'actualité au Gouvernement.

En application de l'article 8 , alinéa 3, de notre règlement, les listes des candidats présentés par les groupes ont été publiées. Ces candidatures seront ratifiées si la présidence ne reçoit pas d'opposition dans le délai d'une heure prévu par notre règlement. L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à la création du Centre national de la musique

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous sommes réunis aujourd'hui pour donner la touche finale à la proposition de loi créant le Centre national de la musique, qui, plus qu'attendu, était espéré par toute la profession depuis 2011, date à laquelle un certain député Franck Riester l'avait évoqué pour la première fois dans un rapport. Il aura fallu attendre que ce député accède à la fonction de ministre de la culture pour que ce véritable serpent de mer englué dans les sables politiques et administratifs voie enfin le jour. Comme quoi, la persévérance et la continuité paient Il a cependant été nécessaire- je tiens à le rappeler -de joindre à vos efforts, monsieur le ministre, ceux de l'Assemblée nationale. La proposition de loi déposée par Pascal Bois et plusieurs députés, elle-même précédée d'un important travail d'analyse mené avec Émilie Cariou, à laquelle je voudrais également rendre hommage, a permis à ce projet de trouver enfin une forme concrète, précise, et de vaincre les scepticismes et les oppositions, et ils furent nombreux. Le Sénat, qui a toujours soutenu la filière musicale et les artistes, notamment du côté de sa commission de la culture, a bien volontiers choisi de jouer le jeu. C'est donc très naturellement que notre commission a travaillé, consciente de la fragilité des équilibres atteints avec la profession, mais déterminée à faire progresser les thèmes qui lui sont chers. Je veux citer comme étant des apports fondamentaux de notre assemblée : l'inscription des notions d'égale dignité des répertoires ainsi que celle, si importante pour nous et notre présidente Catherine Morin-Desailly, de droits culturels au sein même du corpus de règles qui doivent présider au fonctionnement du CNM le renforcement de la mission transversale de développement territorial, en octroyant au CNM la possibilité de conclure des contrats et de nouer des partenariats avec les collectivités territoriales et les acteurs de la filière musicale l'élargissement de la composition du conseil professionnel à l'ensemble des organisations concernées par l'action du CNM, afin de permettre aux collectivités territoriales et aux structures publiques de la musique en régions d'y siéger. Le très large accord recueilli en commission, puis en séance publique au Sénat, sur la proposition de loi permettait d'espérer une commission mixte paritaire conclusive. Celle-ci s'est réunie le 17 septembre dernier, et je suis heureux de dire qu'elle s'est achevée assez rapidement par un accord qui conserve l'intégralité des apports du Sénat. Il semble d'ailleurs, depuis quelque temps, régner en matière culturelle une heureuse convergence de vue entre les deux assemblées. Cela marque, j'en suis intimement persuadé, que, en matière de création et de soutien aux artistes, les députés et les sénateurs sont liés par une vision commune et, surtout, partagée de l'intérêt général. Je suis d'ailleurs heureux de pouvoir souligner la qualité de nos échanges avec Pascal Bois, auteur de la proposition de loi et rapporteur, ainsi qu'avec vous-même et vos services, monsieur le ministre : vous avez contribué à faire de cette proposition de loi de l'Assemblée nationale un texte qui nous rassemble. Maintenant, nous n'allons pas nous contenter d'avoir adopté une belle loi bien écrite. Derrière le texte, il y a la réalité de cette structure à créer et à faire vivre au service de la musique. Il reste encore quelques écueils sur le chemin, et pas des moindres. Premier écueil : la question des moyens, et tout d'abord ceux attribués par l'État. Le projet de loi de finances pour 2020 a levé une partie des doutes, en affectant 7,5 millions d'euros au CNM, auxquels il faut ajouter un demi-million d'euros en provenance du CNV. Sans déflorer un débat budgétaire que nous aurons dans quelques semaines, et qui sera mené par notre rapporteure Françoise Laborde, je tiens, à titre personnel, à exprimer ma satisfaction quant à ce montant, qui correspond à environ un tiers de l'objectif cible de 20 millions d'euros. Cette somme devrait permettre au CNM d'amorcer ses travaux lors de sa première année de fonctionnement. Ainsi, le CNM ne devrait pas passer du statut peu enviable de serpent de mer à celui, encore moins enviable, de coquille vide Ma satisfaction est toutefois tempérée, car je ne trouve nulle trace d'un quelconque engagement pour les années à venir. Et si les mots ont un sens, leur absence est parfois tout aussi éloquente donc, monsieur le ministre, que nous serons vigilants à ce que l'État assume bien sa part au long cours et dans des proportions propres à susciter l'enthousiasme et joue un rôle incitatif à l'égard des financeurs privés. Parlons-en, justement, des opérateurs privés. Certaines craintes ont été émises sur la capacité et la volonté des organismes de gestion collective à abonder le CNM. Le conflit, maintenant porté devant les tribunaux, qui oppose deux d'entre eux- et pas des moindres -pourrait menacer les premiers pas du Centre. Je regrette personnellement ce conflit qui oppose, pour schématiser, « petits producteurs » et « majors au moment même où la maison commune qu'est le CNM se constitue. Sur cette affaire, monsieur le ministre, je serai heureux d'avoir votre sentiment. Après la question des moyens, le second écueil est la participation des professionnels. Nous le savons, tout n'est pas dans la loi. Tout le monde attend avec intérêt- avec angoisse, devrais-je dire -la parution du fameux décret prévu à l'article 2 sur la composition du conseil d'administration et du conseil professionnel. Je sais que les concertations ont d'ores et déjà été lancées, mais il ne faut pas que le délai entre l'accord en CMP et l'adoption définitive du texte accentue la méfiance. En la matière, il vous faudra aller vite au risque de peiner certains, pour ne pas lester de rancoeur la création du CNM. Cette question est d'autant plus sensible que, je le rappelle, les acteurs de la filière musicale sont aujourd'hui globalement majoritaires dans la composition des conseils d'administration des cinq organismes qui devraient disparaître au profit du CNM. Il est absolument essentiel que les différents acteurs de la filière musicale n'aient pas le sentiment d'un marché de dupes en intégrant cette maison commune, faute de quoi le risque serait que certaines des associations de droit privé refusent de rejoindre le CNM, ce qui ferait perdre beaucoup de son intérêt au projet. De même, je vous invite à prendre tout particulièrement en considération la place éminente des collectivités territoriales, qui sont directement intéressées par l'action du Centre. Les défis sont donc nombreux ! Le futur CNM pourra cependant s'appuyer sur la mission confiée à Catherine Ruggeri, qui me paraît tout à fait en ligne avec les ambitions élevées que nous nourrissons, que vous nourrissez, monsieur le ministre, pour le Centre. Catherine Ruggeri effectue un travail remarquable de rassemblement de tous. Je tiens à saluer ici son engagement et à souhaiter que ses compétences ainsi que ses qualités de diplomatie et d'indépendance puissent continuer à bénéficier au secteur. Pour conclure, je voudrais donner les trois orientations qui, selon moi, devraient présider à la naissance du CNM. Première orientation : l'unité. Cette maison doit être celle de toutes les musiques, de tous les musiciens, et ne pas hésiter au passage à aller vers un monde amateur si riche et vivant. Or, comme nous le savons, l'unité est un combat qui suppose, pour être remporté, de l'écoute- d'autant plus en matière musicale -et le respect des autres. J'adresse donc solennellement aux futurs responsables du CNM et à ses grands acteurs un avertissement : le succès sera celui de tous Si échec il y a, il sera lourd de conséquences pour tous, car l'effort que fait aujourd'hui l'État pourrait ne pas se retrouver avant plusieurs longues années. Deuxième orientation : la conscience des défis à venir. Le CNM devra rapidement se saisir des lourds dossiers qui préoccupent la filière musicale. Je veux en citer trois qui me paraissent particulièrement d'actualité. Il s'agit, tout d'abord, de la défense de la conception européenne du droit d'auteur, régulièrement attaquée, pour lui substituer la notion anglo-saxonne de et le partage de la valeur entre les différents intervenants. Le futur projet de loi audiovisuel sera, je pense, l'occasion pour nous de réaffirmer notre vision et, pour le Centre, d'élaborer avec la profession une position commune. ensuite, la concentration dans le secteur de la musique. Sur ce point, qui relève aujourd'hui davantage de l'intuition, nous avons cruellement besoin de données. C'est l'une des raisons pour lesquelles la création du CNM était si importante, car elle devrait enfin permettre le lancement de l'observatoire de l'économie de la musique, prévu par la loi LCAP, mais jamais mis en place depuis. Cet observatoire permettra enfin d'avoir une meilleure connaissance du secteur, une connaissance que je juge indispensable pour définir des politiques publiques plus adaptées, comme le souhaite l'ensemble des acteurs de la filière musicale. N'oublions pas que les questions de concentration agitent aujourd'hui particulièrement le secteur des festivals musicaux. C'est une question urgente si nous voulons préserver le dynamisme de nos festivals, déjà mis à mal par la hausse des coûts de sécurité et des normes en la matière de plus en plus élevées. Enfin, le dernier dossier de cette liste, bien entendu non exhaustive, est l'impact sur la diversité culturelle des algorithmes mis en oeuvre par les services de. Ce dernier point, et le nécessaire dialogue qui devra se nouer avec les plateformes, nécessitera la capacité d'expertise du Centre et son rôle de relais des positions de la filière. Troisième orientation : l'enthousiasme. Au-delà de ce qui vient d'être évoqué, des écueils, des craintes, nous devrions tous nous réjouir sincèrement d'assister à la naissance de ce « CNM à la française », promis à un grand avenir. Cet enthousiasme doit infuser dans le milieu professionnel, qui ne pourra pas dire que l'État, gouvernement et parlement réunis, a été sourd à leurs demandes. Mes chers collègues, vous l'aurez compris, je suis déjà dans « l'après » et dans ces beaux défis que nous abordons avec bonheur, lucidité et détermination.

Les membres de la commission mixte paritaire ont apporté deux clarifications qui assurent une meilleure intelligibilité de la loi. En premier lieu, la disposition qui prévoit un conseil professionnel adjoint au conseil d'administration a été modifiée afin d'éviter une confusion possible avec la notion d'instance représentative du personnel, reconnue en tant que telle par le code du travail. Or, au cas d'espèce, il s'agit bien de faire du conseil professionnel une instance réunissant des représentants des organisations concernées par l'action de l'établissement. En second lieu, il est apparu plus pertinent de mentionner les « données », plutôt que la « donnée », en ce qui concerne l'observatoire du Centre national de la musique. Vous savez combien l'enjeu de la connaissance et de la transparence du secteur est primordial, que ce soit pour mieux comprendre les mutations à l'oeuvre ou bien pour améliorer les dispositifs de soutien ou la régulation du secteur. Le Gouvernement soutient ces modifications. Cet accord témoigne des attentes extrêmement fortes concernant la création d'un établissement public dont la mission principale est de soutenir le secteur de la musique. Le ministre de la culture l'a rappelé ici même devant vous, durant l'examen du texte en première lecture, la création du CNM intervient à un moment crucial pour le secteur de la musique : après la « crise » des années 2000, le retour de la croissance et notamment ses effets pour les créateurs et les entreprises en France ne sont pas acquis de manière définitive. En effet, le marché est mondial, très compétitif et marqué par les rapidités de l'innovation, en particulier la transition numérique. Or la musique est un écosystème fragile en perpétuelle mutation, qui se heurte à certains phénomènes de concentration préoccupants. Le soutien et l'accompagnement de ce secteur par la puissance publique sont donc fondamentaux. Le CNM doit par conséquent contribuer à améliorer et adapter l'action publique en faveur de la musique. La musique est la première pratique culturelle des Françaises et des Français, la deuxième industrie culturelle du pays. L'absence d'un opérateur unique capable de fédérer les acteurs de la musique, d'accompagner et de soutenir les professionnels, d'encourager la création relevait de l'étrangeté. Le texte qui est soumis à votre approbation C'est pourquoi la première de ces adaptations est la création du CNM. Un tel accord a été rendu possible par le dialogue nourri et fécond auquel le texte a donné lieu, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Le Gouvernement se félicite de l'enrichissement du texte, qui a été substantiellement modifié lors de son examen par le Parlement. Outre de nombreuses évolutions rédactionnelles, celui-ci a renforcé les missions et le rôle du CNM, ce qui traduit un sens du dialogue et de l'écoute qu'il convient de souligner. J'en suis témoin sur un autre texte, en cours d'examen ... La responsabilité sociale de l'établissement a été renforcée, que ce soit en faveur de l'environnement et du développement durable, ou encore de l'égalité entre les femmes et les hommes. Le CNM a ainsi désormais pour mission de favoriser un égal accès des femmes et des hommes aux professions musicales. En outre, la parité au sein de ses instances de gouvernance est pleinement consacrée. On ne peut que s'en réjouir collectivement. Par ailleurs, les missions du CNM ont été élargies. Je pense à l'ajout explicite de la création musicale, en faisant référence à la composition, l'interprétation et la production, qui est pleinement conforme à la volonté du ministre de la culture de placer les artistes au coeur du projet du CNM et, plus largement, de l'action gouvernementale en matière de culture. Ce centre devra être consacré au service de l'ensemble de la filière musicale dans toutes ses nuances et tourné vers les créateurs. Les soutiens économiques qu'il mettra en oeuvre seront conçus de manière à promouvoir la diversité culturelle et à favoriser l'innovation. Il placera la dimension territoriale au coeur de son action. Je pense également à la mission de valorisation du patrimoine musical dont les Français sont fiers. Il s'agit là d'un aspect important de la politique culturelle en faveur de la musique, en lien avec les missions de rayonnement et de transmission. Concernant l'enjeu essentiel de la connaissance du secteur et de ses mutations, des avancées notables ont été acquises. On peut ainsi saluer le renforcement des missions d'observation du CNM, que ce soit en matière de recueil des informations utiles- notamment commerciales et financières -et de diffusion de l'information économique et statistique. Enfin, le CNM a été inscrit dans une démarche de concertation permanente, notamment en prévoyant la création d'un conseil professionnel auprès du conseil d'administration. Cette instance de gouvernance est de nature à favoriser le rassemblement, le dialogue et la concertation. Mesdames, messieurs les sénateurs, en adoptant la proposition de loi qui est soumise à votre vote aujourd'hui, vous permettez la création du Centre national de la musique et, avec lui, la mise en oeuvre d'une politique ambitieuse en faveur de la musique. Je n'ignore pas que ce travail de réflexion et de documentation est le fruit d'une concertation avec l'ensemble des acteurs de la filière. Parallèlement à la future loi, une mission de préfiguration travaille activement, en lien avec les structures qui doivent rejoindre le CNM, leurs salariés et les professionnels du secteur- entreprises, organismes de gestion collective, associations, syndicats -, en vue de faire aboutir les chantiers qui assureront le bon fonctionnement de l'établissement.

comprend 7,5 millions d'euros de moyens nouveaux pour lancer le Centre en 2020. Il affecte également au CNM les ressources autrefois dédiées au CNV et aux autres organismes et dispositifs qui ont vocation à rejoindre le nouvel établissement, dont les recettes de la taxe sur les spectacles de variétés,

Edvard Grieg, compositeur et pianiste norvégien, disait que, si les mots ont parfois besoin de musique, la musique, elle, n'a besoin de rien. Nous ferons tout de même oeuvre utile en créant, enfin, une maison commune à la filière musicale, dont le chiffre d'affaires global est supérieur dans notre pays à celui de la filière cinématographique. Le secteur musical, animé par une multitude de chapelles, est aujourd'hui encore profondément éclaté. Dans sa grande sagesse, la Haute Assemblée s'évertue généralement à reconnaître les mérites de chacun. Il convient donc de rendre un légitime hommage à l'implication constante et profonde de M. le ministre de la culture, tout d'abord comme législateur, puis désormais comme membre de l'exécutif, dans l'aboutissement de ce projet. ce dévouement indéfectible à la cause du CNM continuera de l'animer dans les prochaines semaines, lorsque les deux grands « silences » de cette proposition de loi devront faire l'objet de réponses.

comporte tout de même des zones d'ombre significatives sur le fonctionnement du futur établissement public : tout d'abord, en termes de gouvernance ; ensuite, en termes de financement disponible et d'un éventuel abondement de l'État. De ces deux points dépendent très largement la présence et l'engagement des acteurs concernés au sein de la future structure et la réussite du projet. Sans revendiquer l'ambition budgétaire de 100 millions d'euros du premier projet bâti en 2011, dont on connaît le sort funeste, nous souhaitons voir mobilisées des ressources « modernes Le CNM peut en effet légitimement s'appuyer sur des modes de financement innovants, notamment issus du numérique, comme la taxe YouTube ou la taxe Copé. Constitué à partir du futur ex-CNV le 1 janvier prochain, le CNM se verra ensuite consolidé par sa fusion avec l'IRMA- le Centre d'information et de ressources sur les musiques actuelles -, le Bureau export de la musique française, le Fonds pour la création musicale et le Calif, le Club action des labels et des disquaires indépendants français. Même si les cellules constitutives du Centre national de la musique sont plutôt issues du monde des musiques actuelles, le CNM devra être la maison commune de toutes les musiques. Cette structure ne saurait limiter son intérêt aux secteurs marchands les plus pertinents. Il ne s'agit pas d'arroser là où il pleut déjà Profondément affectée par la révolution numérique- la musique enregistrée a vu son chiffre d'affaires divisé par trois entre 2002 et 2015 -, la filière a su se réinventer. Le CNM devra participer de la consolidation de ce nouveau modèle, qu'il soit économique ou productif. Mes chers collègues, attaché à la création d'une maison commune et à la structuration de la filière musicale en France, le groupe du RDSE soutiendra le texte élaboré par la commission mixte paritaire. La parole

paritaire conclusive du 17 septembre dernier de cette proposition de loi ouvrant création du Centre national de la musique est particulièrement bienvenue. Je pourrais dire qu'elle tombe à point s'il n'avait fallu attendre pas moins de huit années pour que ce projet puisse enfin prendre forme. Il faut saluer ici l'opiniâtreté du Gouvernement, en particulier de l'actuel ministre de la culture, Franck Riester, qui a finalement porté sur les fonts baptismaux ce que d'autres, avant, avaient promis, mais n'avaient pu ou su mettre en oeuvre Le Centre national de la musique verra donc le jour le 1 janvier prochain, et ceux qui, il y a encore quelques semaines, émettaient des réserves quant à la volonté de l'État d'y mettre les moyens verront- je l'espère -leur scepticisme viscéral, surtout lorsqu'ils sont dans l'opposition, apaisé par les annonces budgétaires très concrètes contenues dans le projet de loi de finances que nous étudierons très prochainement. Nous réparons, par cet acte, par cette création, une anomalie qui sévissait jusque-là parmi nos instruments, pourtant nombreux, de la politique culturelle de l'État. La musique est en effet de tous les arts notre première muse, notre muse quotidienne ; celle qui fait, comme le chantait Charles Trenet, que « longtemps après que les poètes ont disparu leurs chansons courent encore dans les rues » ... On l'oublie souvent, mais c'est la musique qui fut historiquement la première pierre de l'édifice de toutes les politiques publiques de la culture mises en oeuvre dans notre pays. C'est en effet Louis XIV, « patron des arts qui, tout juste après l'avoir fait naturaliser, nomma le jeune et brillant musicien florentin Jean-Baptiste Lully, en 1661, au titre très exceptionnel de surintendant de la musique du roi. Un véritable ministère de la culture musicale avant l'heure Par la volonté du Roi-Soleil, la musique devenait ainsi plus qu'un simple divertissement privé au service du roi ; elle était désormais élevée au rang d'instrument public de diffusion de la splendeur de son règne, et accessoirement de la France, par l'entremise de la Cour, sur tout le territoire français de l'époque. Pourtant, au fil des siècles, l'État, en France, contrairement à nombre de nos pays voisins, s'est trop peu préoccupé de politique publique en matière de musique. Là où les Allemands, les habitants des ex-pays de l'Est et ceux des pays scandinaves encensent leurs grands compositeurs et favorisent sans limites la pratique amateur de la musique, notre pays a toujours donné la priorité à ses écrivains et à la lecture publique, à ses cinéastes et à la fréquentation des salles. Les politiques en faveur de la musique ont surtout été le fruit de l'attention toute particulière- ce n'est pas le ministre chargé des collectivités territoriales qui me contredira -... Jamais ! ... portée par nos villes et nos collectivités locales. À la différence du cinéma et du livre, qui ont pu, dès 1946, bénéficier de la création quasi concomitante du Centre national de la cinématographie et de la Caisse nationale des lettres, ancêtre du Centre national du livre, il manquait jusqu'à présent une grande institution nationale consacrée à la promotion de la musique et de la chanson sous toutes leurs formes. Je parlais à l'instant des soixante ans du ministère de la culture.

il aura fallu attendre plus de sept ans après la création du ministère pour que celui-ci se dote enfin d'une direction de la musique, confiée à l'excellent compositeur

Pour Marcel Landowski, il s'agissait, d'une part, de « former des musiciens de haut niveau » et, d'autre part, de « rendre l'enseignement musical accessible à tous Cette volonté résonne encore aujourd'hui quand le ministre de l'éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, veut développer l'apprentissage de la musique dans les établissements scolaires en faisant en sorte qu'il y ait des chorales dans toutes les écoles et tous les collèges et en encourageant les pratiques instrumentales. Cette incitation est indispensable, mais si nous voulons que l'industrie musicale française puisse se développer et son poids économique, actuellement estimé à 8,7 milliards d'euros et à quelque 240 000 emplois, augmenter, il est nécessaire qu'elle parle d'une seule voix. Le Centre national de la musique sera cette voix, en regroupant en son sein le CNV, le FCM et l'IRMA.

a pourtant eu bien du mal à s'imposer, qui fait sans doute que nous sommes aujourd'hui presque unanimes pour saluer la création du Centre national de la musique. Alors, ne boudons pas notre plaisir ! C'est pourquoi, monsieur le ministre, mes chers collègues,

orateurs l'ont dit, cela fait maintenant bien des années qu'une large partie des acteurs du secteur réclame la création d'une maison commune de la musique ou, à tout le moins, une clarification des dispositifs existants.

concerne la place du ministère de la culture dans le processus. Celui-ci se met lui-même en retrait de son coeur de mission. S'engager économiquement pour promouvoir le secteur et sécuriser ses professionnels est évidemment une bonne chose, mais, si vous m'y autorisez, monsieur le ministre, signer le chèque ne suffit pas à parler d'engagement ferme dans le secteur de la création. Pour ne prendre qu'un exemple, l'abandon de la mission d'agrément, ouvrant droit à des crédits d'impôt, est préjudiciable et prête le flanc aux mêmes débats sur l'objectivité des aides attribuées En outre, ce désengagement risque d'entraîner une perte du contrôle parlementaire sur les stratégies déployées par le Centre national de la musique. La deuxième réserve tient justement au fonctionnement du CNM, réserve par ailleurs renforcée par les craintes d'une partie des organisations professionnelles d'être exclues ou sous-représentées dans sa gouvernance. Cette question de la représentation a été l'objet de débats en première lecture, mais il me semble que nous n'avons pas encore trouvé de solution parfaitement satisfaisante. La même question se pose d'ailleurs

Les premiers échos que nous avons concernant la stratégie voulue par le comité opérationnel de lancement du CNM interrogent aussi. L'objectif à court terme et la réponse absolue à la crise de la musique seraient le développement du pour l'écoute et les concerts. Il s'agirait donc de reproduire la stratégie du choc qui avait présidé au règlement de la crise de la fin des années soixante-dix, résolue par la généralisation du CD. Il me semble cependant qu'il faut réinterroger ce modèle, qui conduit concrètement à la concentration des moyens de la musique entre les mains de quelques artistes stars en asséchant progressivement le nombre d'artistes et de ventes. Le choix du rend en effet difficile l'émergence de nouveaux artistes. Il crée en outre une dépendance vis-à-vis de plateformes qui restent financièrement instables et qui généralisent un modèle de rémunération extrêmement faible des artistes, en éliminant

et affaiblit plus généralement les artistes éloignés du monde des musiques actuelles. Notre troisième réserve concerne évidemment- vous n'en serez pas surpris, et d'autres

En termes d'apport de l'État, le montant de 20 millions d'euros avancé par notre commission ne sera pas au rendez-vous, puisque le projet de loi de finances prévoit des chiffres très différents qui nous inquiètent. On doit en effet s'attendre à ce que le CNM ne soit pas pleinement opérationnel dès comme nous le croyons, il bénéficie d'un apport de moins de 8 millions d'euros, ce qui est beaucoup trop faible pour permettre un démarrage correct. Pourtant, le recrutement d'agents pour arriver à 111 personnes, contre 35 au CNV, augurait augurait d'une ambition bienvenue. J'espère que nos craintes seront apaisées et, surtout, que les professionnels du secteur et les élus locaux seront rassurés. Comme je le disais en préambule, au regard de l'urgence, nous voterons

d'ici à quelques mois, le Centre national de la musique verra le jour, fédérant l'ensemble des acteurs de la filière musicale française. Je me réjouis de l'écoute du Gouvernement, en particulier du ministre de la culture et de son implication dans ce dossier. La commission mixte paritaire s'est mise d'accord sur un texte volontairement général. La gouvernance de l'établissement sera précisée par décret, et son financement de 50 millions d'euros sera prévu par le prochain Il s'agit d'accompagner à la fois le développement des forces institutionnelles, des lieux de musique et le rayonnement des artistes, qui interprètent et enrichissent un vaste répertoire, classique ou moderne. Il s'agit aussi de promouvoir toutes les formes de musique, dont la chanson française, qui n'est pas assez mise en valeur. Elles constituent un patrimoine musical dont nous pouvons être fiers Cette première sphère d'artistes et de créateurs est accompagnée de maisons de disque, de journalistes, de professeurs, d'ingénieurs du son, de luthiers, de facteurs de pianos et d'orgues, sans lesquels aucun disque, aucune représentation, ne pourrait voir le jour. La diversité et la complémentarité entre les structures permettront à chaque musicien de trouver les ressources dont il a besoin pour développer sa carrière. Il s'agit, aussi, de réduire les fractures géographiques, sociales, culturelles au travers de la diffusion de la musique, sous toutes ses formes, sur l'ensemble du territoire.

Le « plan de dix ans » élaboré par André Malraux a permis la création d'un réseau d'institutions décentralisées poursuivant cet objectif de rendre la musique accessible à tous. Jack Lang a poursuivi cette politique de démocratisation. Aujourd'hui, pas une région n'est sans orchestre, sans festival, sans salle de concert. La vitalité de la scène musicale exerce une force d'attraction sur les plus grands artistes étrangers. Les services culturels des ambassades sont une vitrine de la création musicale française. Je prendrai l'exemple l'année culturelle France-Égypte, lancée à l'opéra du Caire en début d'année. Autre exemple : La Folle journée de Nantes, qui accueille plus de 130 000 visiteurs chaque année, s'est exportée en Espagne, au Japon, en Russie. La politique des quotas de diffusion, renforcée en juillet 2016, est une réussite. Un renouveau de la politique musicale s'est manifesté avec l'ouverture de la philharmonie de Paris en 2015 et la signature d'un protocole d'accord pour un développement équitable de la musique en ligne. La filière reste fragile, malgré une récente reprise de la croissance du secteur de la production musicale. Le représente désormais plus de 50 % des ventes globales ... L'accompagnement de la numérisation de la filière est un enjeu majeur pour assurer la compétitivité de l'économie de la musique à l'échelle mondiale. C'est une mission essentielle du futur Centre national de la musique.

du projet de loi de finances pour 2020, notre groupe soutiendra le financement du Centre national de la musique tel qu'annoncé par le ministre de la culture, ainsi que la préservation du crédit d'impôt en faveur de la production Enfin, le projet de loi sur l'audiovisuel est très attendu par les acteurs de la filière, avec notamment le renforcement de la lutte contre le piratage. Monsieur le ministre, mes chers collègues, l'ouverture de la culture au plus grand nombre reste au coeur des préoccupations qui animent la rue de Valois et le Sénat.

Mes chers collègues, je suis heureux de saluer en votre nom la présence, dans notre tribune d'honneur, d'une délégation de l'Assemblée nationale d'Arménie, conduite par M. Vladimir Vardanyan, président du groupe d'amitié Arménie-France, président de la commission des lois. Elle est accompagnée par notre collègue Gilbert-Luc Devinaz, président du groupe d'amitié France-Arménie. Cette visite s'inscrit dans le cadre des échanges interparlementaires approfondis entre nos deux assemblées. Elle intervient alors que l'Arménie est engagée dans un vaste champ de réformes, notamment dans le domaine de la justice. Outre des entretiens organisés au Sénat, la délégation se déplacera pour rencontrer des élus locaux et divers spécialistes de l'aménagement local. Nous souhaitons à nos amis arméniens un séjour et des échanges fructueux, en formulant le voeu que cette visite réponde utilement à leurs préoccupations. Nous leur souhaitons la bienvenue au Sénat français

Les deux assemblées sont logiquement parvenues à s'accorder sur ce texte, qui est resté un projet pendant plus de huit ans. La musique va enfin avoir sa maison commune ! Dans l'idéal, le CNM a vocation à fédérer les structures de la filière afin de soutenir les professionnels du secteur musical sur l'ensemble de la chaîne Il doit répondre aux attentes de la filière et être un outil efficace, une instance de dialogue et de cohésion entre les acteurs du secteur de la musique et des variétés dans un contexte de révolution numérique. Il aidera aussi à porter notre musique dans le monde demain, mieux qu'aujourd'hui en tout cas. Il sera aussi un lieu d'observation privilégié qui nous fait aujourd'hui cruellement défaut. Bref, il devra apporter de l'harmonie à ce qui représente actuellement la première pratique culturelle des Français et la deuxième industrie culturelle de notre pays. En effet, le monde de la musique avait face à lui de nombreux organismes- cinq principalement. Leur séparation nuisait à la lisibilité de nos politiques publiques, était source de complexité pour les professionnels et limitait les interactions créatrices entre des secteurs jusqu'à présent artificiellement séparés. Cependant, Cependant, la fusion en une seule et unique instance ne doit pas être synonyme de concentration- nous l'avons dit en première lecture -, alors que les inégalités culturelles sont nombreuses, trop nombreuses, en France. C'est ainsi que, toujours dans un cadre idéal, l'accompagnement des initiatives locales et des collectivités territoriales devra être renforcé par l'intermédiaire du CNM, afin de garantir les droits culturels. Le Sénat a d'ailleurs substantiellement enrichi la proposition de loi de l'Assemblée nationale, en particulier avec l'inscription de l'égale dignité des répertoires et des droits culturels comme principes de fonctionnement du CNM. Ainsi, le ton est donné le Centre aura pour mission d'assurer le respect des droits culturels, la liberté et la diversité de l'expression musicale ainsi que de ses acteurs, professionnels comme amateurs et leur intégrale accessibilité.

qui ne présentent pas seulement des. Tous les territoires et tous les genres musicaux doivent avoir leur place au sein du Centre national de la musique, et c'est ce à quoi nous avons veillé avec notre

Diversité sur le territoire, diversité des acteurs et diversité culturelle : c'est uniquement avec cette volonté que le CNM pourra devenir une véritable « maison commune de la musique » bien orchestrée. Je souhaite cependant, de nouveau, appeler votre attention sur la problématique du financement de ce nouveau centre national. Les documents budgétaires rendus publics par le ministère prévoient que 7,5 millions d'euros seront mobilisés l'an prochain sur le programme 334, sommes qui viendront s'ajouter aux moyens publics déjà consacrés au secteur. : nous voyons bien que nous sommes encore loin de la somme de 20 millions d'euros supplémentaires nécessaires au nouveau centre pour la bonne conduite de ses missions, telle que préconisée par le rapport Bois-Cariou et sur laquelle s'accordent l'ensemble des acteurs. Nous touchons là la corde sensible du projet. Nous serons donc très vigilants sur ce point lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2020. Les modalités de l'administration des crédits d'impôt en faveur de la production phonographique et du spectacle vivant ne me paraissent pas non plus tout à fait résolues,

Enfin, je veux saluer le travail effectué par notre chambre pour renforcer la mission transversale de développement territorial du CNM, en lui octroyant la capacité de conclure des contrats et de nouer des partenariats avec les collectivités territoriales et les acteurs de la filière musicale. Renforcer les actions de développement dans les territoires marque une véritable avancée. Dans la même mesure, conformément au voeu du Sénat, nous souhaitons élargir la composition du conseil professionnel

Monsieur le ministre, je vous laisse dire à votre collègue de la culture, qui, je le sais, y est particulièrement attentif, que la création du Centre national de la musique est une avancée importante pour la vitalité culturelle, et pas uniquement musicale, Nous lui sommes reconnaissants d'avoir ainsi porté, avec tant d'autres, ce projet, de l'avoir mené à la baguette, d'abord comme député puis aujourd'hui comme ministre. Il reste cependant encore du chemin à parcourir pour que cette structure soit pleinement efficiente. C'est pourquoi nous n'irons pas plus vite que la musique : la mise en place effective du CNM dans les mois qui viendront fera l'objet de toute notre vigilance. Nous avancerons pas à pas

Robert. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, « enfin ! », serais-je tentée de dire ... Après une décennie à esquisser les ébauches d'une maison commune de la musique, ses fondations sortent finalement de terre. Il reste des questionnements substantiels à régler, en particulier son financement et sa gouvernance, mais nous aurons l'occasion d'en débattre prochainement. réjouissons-nous que tous les acteurs de la filière, dans leur entière diversité, puissent échanger, partager leurs analyses et réfléchir collectivement aux mutations constantes qui traversent le secteur au sein d'un même forum. Au regard des changements qui bouleversent le monde de la musique, établir un espace de dialogue commun était devenu impérieux. Dès lors, le Sénat a pleinement oeuvré à ce projet. D'ailleurs, presque la totalité des apports validés en première lecture ont été confirmés au cours de la commission mixte paritaire. Je voudrais remercier notre rapporteur, qui, dans un esprit constructif, a effectué un important travail et a permis de dégager une unanimité autour de cette proposition de loi. Ainsi, le texte a été enrichi à de multiples endroits. Je ne ferai pas une liste à la Prévert, mais j'aimerais néanmoins insister sur plusieurs points. En premier lieu, dans la continuité de la loi NOTRe et de la loi LCAP, la mention des droits culturels et le renvoi à la convention de l'ONU me paraissent fondamentaux. Outre l'accent mis sur la promotion de la diversité culturelle, il s'agit aussi de reconnaître le rôle émancipateur de la musique par la pratique et la participation de toutes et tous à la sphère musicale. lieu, il était inconcevable que l'artiste soit complètement invisible dans cette proposition de loi. Au travers du « soutien à l'écriture, à la composition et à l'interprétation », qui figure désormais à l'alinéa 4 de l'article 1, nous revenons aux sources de la création et marquons notre profond attachement aux auteurs, compositeurs et interprètes sans qui nulle création musicale ne serait possible. Vous savez que, à titre personnel, j'aurais aimé aller plus loin, en proposant une expérimentation, un fonds de soutien. cela se fera plus tard. Enfin, le numérique impactant massivement le secteur musical, la prise en compte des usages et de la valeur de la donnée est essentielle. la mission de l'observatoire de l'économie sera décisive, car elle favorisera l'innovation et l'adaptation permanente des acteurs aux mutations socio-économiques, mais aussi aux comportements des usagers. usagers. Maintenant que le CNM devient réalité, plusieurs paramètres me semblent cardinaux afin de garantir sa réussite. Tout d'abord, sa représentativité, à tous niveaux, doit être assurée. Je pense singulièrement au conseil professionnel, « instance réunissant des représentants des organisations directement concernées

doit témoigner de la diversité du secteur. En parallèle, la représentativité fait écho à la pluralité des esthétiques, soulignée par la très belle expression d'« égale dignité des répertoires » qui composeront nécessairement le futur CNM. ailleurs, comme je l'ai spécifié précédemment, je crois que les missions du CNM doivent dépasser les attributions originelles du CNV, sous peine de manquer le changement d'envergure que nous prônons collectivement. collectivement. Par-delà la fonction de soutien financier au secteur musical, des préoccupations « d'intérêt général » devraient l'animer- d'ailleurs, cette conception se reflète dans ses missions. Sans aucunement se substituer à l'action menée par le ministère de la culture, le CNM n'en demeure pas moins une enceinte où l'État sera majoritaire et garant de cette mission de service public. Par conséquent, nous attendons de l'État qu'il joue un rôle actif, qu'il soit force de propositions à destination de la filière, mais aussi très mobilisateur sur les dossiers épineux du moment et stratège sur les grands enjeux. le CNM sera ce que les acteurs du secteur décideront d'en faire. Ces derniers se l'approprieront, établiront leurs priorités, feront émerger des problématiques nouvelles et renforceront probablement son action sur certaines questions majeures. Je pense au soutien à la diversité musicale, à l'émergence de nouveaux artistes, au partage de la valeur, à la mise en oeuvre du pass culture, à l'égalité entre les femmes et les hommes ou encore à la formation professionnelle. En outre, la place et le positionnement du CNM seront déterminés par les coopérations qu'il entendra mener avec ses différents partenaires. ouvertes par l'alinéa 15 de l'article 1, qui dispose qu'il « associe les collectivités territoriales et leurs groupements à l'exercice de ses missions », soient le plus larges possible. La possibilité de conclure des contrats et de nouer des partenariats avec les collectivités est un formidable levier pour conférer un ancrage territorial au CNM. Au final, la concrétisation du CNM arrive à point nommé. Nombreux sont les chantiers qui l'attendent. J'en citerai quelques-uns, le soutien public à la production et à la création musicales, à travers la pérennisation et la montée en charge des crédits d'impôt production phonographique et spectacle vivant.

finir, j'évoquerai un problème vital- M. le rapporteur l'a déjà abordé -, qui me tient à coeur : le phénomène de concentration dans le secteur musical. Si nous en percevons nettement les contours, si nous en pressentons l'emprise, nous avons encore besoin de l'objectiver. Nous avons besoin de comprendre ses origines et ses ramifications. les instruments d'une éventuelle régulation par la puissance publique, à laquelle pourraient prendre part les acteurs de la filière, afin d'éviter tout abus de position dominante et en vue de contrecarrer les effets pervers qui se font déjà sentir en termes de diversité musicale. Monsieur le ministre, mes chers collègues, au fond, ce qui est implicitement en jeu, c'est une forme d'identité culturelle revendiquée par la France dans le monde, une « marque de fabrique dans la droite ligne de notre exception culturelle, si je puis m'exprimer ainsi. Je ne doute pas que le CNM sera de cette bataille, porteur, pour paraphraser le titre d'un célèbre roman de Romain Gary, de sa propre « promesse de l'aube ».

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je me réjouis que l'idée d'une maison commune de soutien à la création musicale, véritable serpent de mer de la politique culturelle française, puisse enfin se concrétiser dans le texte que nous allons adopter aujourd'hui. En effet, si la musique est la première pratique culturelle et la deuxième industrie culturelle dans notre pays, elle sera la dernière filière artistique à disposer d'un centre national. Je rappelle que le projet a été lancé par le Président Sarkozy, à l'issue d'une mission dont l'actuel ministre de la culture était le rapporteur, au moment où l'industrie musicale traversait le plus fort d'une crise liée aux nouveaux modes d'écoute, au développement du et au piratage de masse. L'alerte était lancée alors que le chiffre d'affaires de la On comprend donc l'inquiétude qui fut celle des acteurs concernés lorsque le projet a été délaissé sous le quinquennat de François Hollande. Depuis, l'industrie musicale connaît un nouvel essor. Les acteurs français ont finalement su tirer parti du et la fréquentation des concerts a augmenté. cet équilibre reste fragile. La crise a bien montré le danger, pour l'industrie musicale, de demeurer une filière morcelée. Il est aujourd'hui essentiel que celle-ci puisse défendre ses intérêts collectifs, dans une stratégie de long terme. À cet égard, ce texte est particulièrement attendu. Le Centre national de la musique jouera un rôle important d'observation du fonctionnement de la filière, afin de déterminer les actions politiques à mener. Il pourra justifier auprès de l'administration l'impact de concours financiers bien souvent remis en cause. Son rôle sera majeur en matière de diversité culturelle. Je me réjouis que la Haute Assemblée ait pu préciser et élargir ses missions lors de l'examen de la proposition de loi. Je citerai notamment le rôle du CNM dans la collecte d'informations économiques et statistiques au sein de la filière musicale, le soutien qu'il apportera à l'exportation des productions françaises et à la mobilité des artistes l'introduction du « respect de l'égale dignité des répertoires ». Surtout, en tant que représentants des territoires, nous nous sommes attachés à mieux reconnaître la place des collectivités dans la mise en oeuvre de la politique musicale il est mentionné expressément qu'elles pourront conclure des contrats et nouer des partenariats avec le CNM et qu'elles seront associées au comité professionnel. Je tiens à remercier le rapporteur Jean-Raymond Hugonet de son travail constructif et de son investissement personnel proposition de loi. Un texte commun ayant été élaboré avec l'Assemblée nationale, le CNM devrait être juridiquement fonctionnel au 1 janvier 2020. Il restera cependant plusieurs points à préciser pour l'avenir : d'abord, la gouvernance du Centre national, qui sera définie dans un décret statutaire, en cours de préparation, dont nous souhaitons qu'il respecte la présence des différents acteurs de la filière ensuite, le budget alloué au CNM pour mener à bien ses missions, qui devra comporter des moyens nouveaux. Je rappelle que ceux-ci ont été estimés par la mission de préfiguration à 20 millions d'euros en année pleine. je m'associe aux préoccupations exprimées par notre rapporteur concernant la somme de 7,5 millions d'euros qui a été annoncée pour 2020. Le CNM sera le fer de lance et la vigie de la diversité musicale. Encore faut-il qu'on lui en accorde les moyens Je veux, pour terminer, évoquer la question du piratage. Si une enquête de la Fédération internationale de l'industrie phonographique a relevé une progression de la consommation de musique, 27 % des consommateurs utilisent des moyens frauduleux. L'écosystème illicite se complexifie, avec l'apparition d'une pluralité d'acteurs intervenant en amont ou en aval des pratiques de piratage pour mieux les organiser et le perfectionnement des mesures de contournement. Dans ce contexte, il faut revoir notre système de protection. J'espère que nous aurons prochainement des précisions sur les mesures envisagées par le Gouvernement, puisqu'une fusion du CSA et de la Hadopi a été annoncée dans le cadre de la réforme de l'audiovisuel, sans que nous connaissions les aménagements que cette décision induira pour la protection des droits d'auteur. La musique est un secteur particulièrement soumis aux évolutions technologiques. Dans ce contexte, le législateur doit savoir adapter rapidement notre droit. La présente La présente proposition de loi contribuera à garantir l'équilibre de la filière. En dehors des points de vigilance que j'ai indiqués, les membres de notre groupe adhèrent bien évidemment aux dispositions de ce texte et lui apporteront tout leur soutien. La discussion

la mise en place du conseil d'administration et du conseil professionnel, mais aussi, et surtout, le vote de la loi de finances, car d'aucuns craignent que ce nouvel outil ne soit qu'une coquille vide. Nous aurons, mes chers collègues, à veiller de manière très précise et très concrète

dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, l'ensemble

que nous puissions conforter l'engagement citoyen des personnes handicapées à l'approche des élections municipales, en leur évitant l'application de la regrettable interprétation

d'humanité où nous traitons de l'une de nos valeurs, l'égalité de tous les citoyens. Monsieur le ministre, moi non plus, je ne vous ferai pas de procès d'intention. Nous avons eu l'occasion

alors que, le Gouvernement comme nous tous, nous nous inquiétons pour 2020 d'un manque de volontaires pour prendre des responsabilités, souvent dans nos petites communes, cette loi, qui s'appelle Engagement, est l'occasion de donner la chance à tous les citoyens qui le souhaitent de pouvoir jouer un rôle important dans la cité. « Par ailleurs, quelle place veut-on donner aux personnes handicapées ? Elles ont toute leur place parmi nous. » Je vous remercie, monsieur le ministre, d'oeuvrer pour que nous trouvions avant la fin de nos débats

l'ancien Président de la République Jacques Chirac, à qui nous avons rendu hommage, prononçait ces mots au sommet de la Terre à Johannesburg. Dix-sept ans après, les Français mesurent tous tous l'importance du défi environnemental. Il est de notre responsabilité, dans cette assemblée, de nous préoccuper de la terre que nous voulons transmettre à nos enfants et aux générations futures. En la matière, nous avons beaucoup à attendre des chefs

C'est pourquoi cet amendement vise à autoriser le maire à édicter des mesures spéciales destinées à limiter les nuisances environnementales générées par la circulation des véhicules ainsi que par les navires mouillant dans les baies maritimes. Quel est l'avis de la commission

nous ne laisserons pas sortir le texte du Sénat sans que ce problème ait été résolu. Vous demandez la confiance à l'égard du Gouvernement. Je demande la confiance à l'égard du Sénat. En d'autres termes, si vous n'êtes pas sûr que notre amendement remplisse toutes les conditions pour être validé, nous préférons néanmoins qu'il soit adopté et transmis à l'Assemblée nationale, ce qui vous laissera largement le délai nécessaire pour lever tous les tous les éventuels inconvénients que vous redoutez. Il me paraît très important que, à défaut d'une réponse du Gouvernement sur le fond

Monsieur le président de la commission des lois, je me suis engagé devant vous, avant même que ce texte ne débute, à m'inspirer des travaux du Sénat et à faire acte de coproduction.

nombre d'interventions, j'ai complètement changé les avis du Gouvernement, parce que nous étions sur une matière dont j'étais le chef de file politique et que le Président de la République et le Premier ministre m'ont confié la responsabilité des collectivités territoriales. En tant que chef de mon administration, de donner la parole du Gouvernement sur des sujets liés à l'intercommunalité, au code général des collectivités territoriales. Or nous parlons là d'une matière à la fois sociale et fiscale. D'ailleurs, c'est bien pour cela que la Constitution et les règlements des assemblées

Boissy-l'Aillerie, ville située dans le département de Rachid Temal, qui est à l'origine de cet amendement, ce sont 4 500 mètres cubes de déchets ménagers et gravats qui ont dû être retirés. La remise en état du terrain agricole aura coûté pas moins de 320 000 euros à la commune. cet amendement, il est proposé de faire le choix de la sécurité juridique pour les maires qui font déjà un usage répressif de la vidéoprotection au titre de la protection des bâtiments et installations publics et leurs abords.

un dispositif totalement similaire a été voté dans le projet de loi Économie circulaire, et nous ne souhaitons pas que cet amendement vienne

nous ne souhaitons pas faire de ce texte un moyen de consacrer des mesures trop répressives, dont l'efficacité reste douteuse, et qui ajoutent bien des responsabilités sur le dos des élus locaux.

que la question de l'astreinte ou de l'amende soit systématiquement interprétée comme une volonté abusive de la part du Sénat

d'une bande de terrain afin d'y effectuer un certain nombre d'aménagements, le plus souvent d'ordre sécuritaire. Cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel, non pour la disposition en elle-même, mais au motif que le législateur a méconnu sa propre compétence. Il apparaît opportun d'autoriser à nouveau cette facilité bien connue et appréciée des élus. Elle permet de libérer du foncier pour réaliser les travaux d'aménagement d'une voirie dans un lotissement sans pour autant

du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social, puis supprimée par l'Assemblée nationale.

avec les moyens dont nous disposons, en particulier les moyens numériques et ceux que nous offre internet pour accélérer les procédures,

Aujourd'hui, une commune qui met en place sur son territoire un dispositif de vidéosurveillance mandate un officier habilité à exercer ce rôle de surveillance. Chaque commune peut effectuer cette démarche, mais il n'y a pas de possibilité de mutualisation des agents et des équipements. Par cet amendement, une personne habilitée sur une commune à assurer la surveillance pourrait le faire pour le compte d'autres communes dès lors que les élus le décideraient, par convention ou par mandat.

de la délinquance, les groupements de communes peuvent ainsi mettre en oeuvre des systèmes de vidéoprotection et les mettre à disposition de leurs communes membres. Par ailleurs, comme le rappelle une circulaire du ministre de l'intérieur du 12 mars 2009,

consultation est alors lancée, qui fait l'objet d'un affichage sur les lieux du projet et dans les mairies des communes dont le territoire est censé être affecté. C'est le plus souvent de cette façon que nos maires sont informés. Ce n'est pas normal

L'amendement a été rectifié en lien avec la commission des lois. Il vise donc finalement à prévoir que le maire doit être informé lorsqu'une demande d'autorisation de défrichement est déposée auprès de l'autorité compétente de l'État par l'un des administrés de sa commune. Ce droit s'exercerait avant que l'autorisation ne soit octroyée, puisque la notification au maire interviendrait à la réception par l'autorité compétente de la demande d'autorisation, et non à l'issue de son instruction, comme c'est le cas aujourd'hui. Quel

par la commission des lois visent à donner de nouveaux pouvoirs ou de nouvelles facultés aux élus locaux, notamment pour réglementer différents dispositifs en matière d'occupation et d'encombrement du domaine public. À ce titre, je souhaiterais formuler deux remarques. le dispositif de l'article 15 ne puisse pas s'appliquer aux établissements publics territoriaux, l'article L. 512-2 du code de la sécurité intérieure permettant aux établissements publics de coopération intercommunale

ils ne peuvent pas le faire appliquer, en raison de l'absence d'agents compétents pour constater et réprimer les infractions aux dispositions des articles R. 632-1, R. 633-6, R. 635-8 et R. 644-2 du code pénal.

je suggère au Gouvernement d'étendre par la voie réglementaire les pouvoirs des agents de surveillance de la voie publique, les ASVP, au constat et à la verbalisation des infractions d'abandon de déchets ou de matériaux. Cette possibilité existe déjà pour les gardes champêtres et les agents de surveillance de Paris. Pourquoi ne pas la donner aux ASVP, qui sont déjà agréés par le procureur de la République pour constater, en application des dispositions de l'article L. 130-4 du code de la route ou de l'article L. 1312-1 du code de la santé publique, certaines contraventions tant au code de la route qu'à la propreté de l'espace public

Dans le cadre de l'exercice de leurs pouvoirs de police, les maires se trouvent souvent démunis pour sanctionner le non-respect de la réglementation. de la réglementation. La voie pénale n'est pas toujours adaptée, notamment en raison des classements sans suite, et n'apporte aucune solution pour la réparation des dommages. Or, dans le cas des manquements aux pouvoirs de police du maire, il est nécessaire d'intervenir assez rapidement,

la condition selon laquelle le comportement doit être répétitif ou continu, et complète le mécanisme de l'amende administrative par celui des astreintes et de l'exécution d'office, aux frais du contrevenant. Concernant l'exécution d'office, plutôt que d'opter pour la consignation d'une somme entre les mains du comptable public avant l'exécution d'office, l'amendement prévoit que les travaux soient réalisés et que la somme soit ensuite réclamée aux contrevenants.

Il nous paraît tout d'abord disproportionné de supprimer la condition relative au risque pour la sécurité des personnes, qui reste un élément essentiel et permet de limiter la procédure de l'amende aux manquements les plus graves. Par ailleurs, l'ajout d'une procédure d'astreinte et d'exécution d'office n'apparaît pas utile en l'espèce, car le maire dispose d'un pouvoir d'exécution d'office en matière d'élagage et de dépôts sauvages. C'est pourquoi la commission formule une demande de retrait. À défaut, l'avis serait défavorable.

lois, de la possibilité pour le maire de sanctionner par des amendes des manquements aux arrêtés municipaux. Nous proposons de prévoir que les manquements aux arrêtés du maire visés par le présent article devront avoir un caractère répétitif et continu pour pouvoir être sanctionnés par une amende administrative. En effet, s'il nous paraît légitime de donner au maire des outils plus efficaces pour faire respecter les arrêtés pris en vertu de ses pouvoirs de police, il nous semble nécessaire d'encadrer cette nouvelle possibilité afin de limiter et de proportionner son caractère répressif. L'amendement

par exemple sur le trottoir ou dans un square, ou qui stockent leurs biens dans un recoin ou les transportent dans un chariot. Au passage, je rappelle qu'aujourd'hui nous n'avons pas suffisamment d'hébergements d'urgence.

imposées par un arrêté est de nature à créer un risque pour la sécurité des personnes. Il s'agit d'un enjeu de tranquillité publique. En outre, le fait de contrevenir à la réglementation, y compris municipale, en matière de vente d'alcool peut d'ores et déjà être puni par une amende forfaitaire. Cela garantit

Les dispositions légales générales applicables aux décisions administratives prévoient que le principe du contradictoire doit pouvoir s'exercer soit de manière écrite, soit de manière orale. C'est le cas pour toutes les mesures de sanction administrative. Il n'y a pas ici de raison d'introduire une exception. Par ailleurs, dans la mesure où l'amende administrative constitue une décision ayant valeur de sanction, il convient de lui appliquer les principes du droit pénal, notamment en matière de droits de la défense. Dans ce contexte, limiter les conditions du contradictoire

ce délai passé, le maire met en demeure le contrevenant qui doit se conformer dans un nouveau délai de quinze jours. Ainsi, si un individu ne prête pas attention aux demandes du maire, il pourra se passer un mois avant que l'amende ne lui soit infligée. Cet amendement vise donc à réduire chacun de ces deux délais

Partout en France, ces élus éprouvent le même sentiment de ras-le-bol face à la multiplication des incivilités et des agressions verbales ou physiques dont ils font l'objet dans l'exercice de leur mandat. Les maires, premiers représentants de l'État dans nos communes, doivent être mieux protégés dans leurs fonctions, tout particulièrement dans les territoires ruraux. En tant qu'officier de police judiciaire, un maire ou un adjoint au maire peut disposer d'un carnet à souche d'amendes forfaitaires, afin de verbaliser lui-même les contraventions susceptibles d'être sanctionnées par le système de l'amende forfaitaire. Toutefois, les maires sont impuissants lorsqu'il s'agit de réprimer des infractions ne relevant pas de la simple contravention auxquelles ils sont pourtant directement confrontés ou dont ils sont les victimes : violences physiques, violences verbales, outrages, destruction, dégradation ou détérioration de biens appartenant au domaine public mobilier ou immobilier.

Il y a un décalage entre l'arsenal théoriquement très répressif et une réponse pénale concrètement peu dissuasive, qui ne permet pas d'enrayer la progression des incivilités.

La mise en place d'amendes forfaitaires délictuelles permet une réponse plus rapide, plus effective, donc plus dissuasive. Quel

ces sanctions sont rarement appliquées. Pour plus d'efficacité, il est proposé d'instituer un système d'amendes civiles en matière de publicité sauvage sur le mobilier urbain et sur le sol. Prononcée par le préfet, l'amende civile pourrait, par son coût plus élevé, avoir un caractère plus dissuasif que le dispositif actuel.

aujourd'hui limité à certains contentieux dans lesquels les fautes commises sont très lucratives, principalement en matière de pratiques restrictives de concurrence et d'atteinte au droit de la propriété incorporelle. L'extension de l'amende civile

de plus en plus confrontés à ce type d'incivilités, qui portent non seulement atteinte à l'environnement, mais pèsent également lourdement sur les budgets des collectivités locales. Le présent amendement vise à autoriser les maires et les adjoints, qui ont la qualité d'officier de police judiciaire, conformément à l'article 16 du code de procédure pénale, à faire procéder, après autorisation du procureur de la République, à l'immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule ayant servi à transporter les déchets, matériaux et autres objets abandonnés, jetés ou déversés illégalement.

la route permettent aux officiers de police judiciaire et aux agents de police judiciaire d'immobiliser et de mettre en fourrière, après accord du procureur, un véhicule ayant servi à réaliser